et le soir : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

des décisions qu'elle a fait adopter ont été annulées par le tribunal administratif. À ce sujet, je tiens à rassurer Laure Darcos, tout le monde a très bien supporté cette épreuve ! Mme Pécresse a fait appel

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

vise à supprimer le présent article, qui fige dans la loi le périmètre dans lequel un étranger ayant franchi la frontière intérieure du territoire national pourra faire l'objet d'une décision de refus d'entrée et non pas d'une décision d'éloignement. Aujourd'hui, si un étranger

de la personne concernée, tant devant le juge administratif que devant le juge des libertés et de la détention lorsque ceux-ci sont saisis dans le cadre de procédures de maintien en zone d'attente. Cela a été dit, la généralisation de la vidéo-audience est particulièrement problématique dans le cadre du droit d'asile et du droit des étrangers, car l'oralité revêt une dimension majeure pour la compréhension par le juge du parcours de la personne étrangère. Outre les difficultés pratiques rencontrées, cette technique déshumanise les débats et ne permet pas d'échanger dans de bonnes conditions. Elle crée une distance préjudiciable aux droits de la défense. En outre- cela a été évoqué lors de la défense de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité -, l'élargissement du recours à la visioconférence sans le consentement de l'étranger contrevient au droit à un procès juste et équitable et présente des risques d'inconstitutionnalité. À cet égard, le Défenseur des droits relève que la mise en oeuvre de la vidéo-audience, contrairement aux exigences liées au droit à un procès équitable, affecte notamment la publicité des débats, le respect du contradictoire et les droits de la défense- comme dirait l'autre, « je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même ». Sur ce dernier point, la garantie des droits de la défense implique la mise en oeuvre d'un dispositif permettant la préparation des débats entre

Sur ce dernier point, la garantie des droits de la défense implique la mise en oeuvre d'un dispositif permettant la préparation des débats entre les avocats et leurs clients en amont de l'audience avec l'assistance d'un interprète et avec des garanties de confidentialité. Aussi des locaux adaptés à la présence physique d'un avocat et d'un interprète aux côtés de l'étranger apparaissent-ils nécessaires avant et pendant l'audience. Enfin, dans le cadre des appels formés contre les ordonnances de maintien en zone d'attente prises par le juge des libertés et de la détention, l'article 10 prévoit que le juge pourra rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée sans avoir préalablement convoqué les parties. Cette disposition porte atteinte au droit à un recours effectif et à l'accès au juge, en violation de l'article 47 de la Charte de l'Union européenne, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». Pour toutes ces raisons, nous demandons que les dispositions de cet article soient supprimées.

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 de l'article 10 du projet de loi. Cet article généralise le recours à l'audience par visioconférence, et ce même sans l'accord du requérant

salle d'audience relevant du ministère de la justice et non du ministère de l'intérieur, audition de l'intéressé ou de son conseil, concours d'un interprète et communication du dossier. Enfin, le traitement par ordonnance dite de « tri » des appels irrecevables existe déjà pour la rétention administrative. L'avis de la commission est

M. Didier Marie. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéoconférence sans l'accord du requérant depuis la salle de la zone d'attente en cas de recours contre une décision de refus d'entrée. La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le tribunal administratif compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle, qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d'organisation des audiences. Or on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques. Une audience se tenant par vidéoconférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéoconférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure,

Le scrutin est ouvert.

du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention et, éventuellement, pour demander que cet appel soit suspensif. Toutefois, la pertinence de cette mesure adoptée par commission des lois n'a pas fait l'objet d'une évaluation approfondie. Cet allongement est justifié par la même logique que celle qui a été appliquée aux articles 16 et 17 concernant les personnes placées en centre de rétention administrative, et non en zone d'attente. Or ces deux situations ne sont pas comparables. Le nombre de personnes placées en centre de rétention administrative chaque année, et par conséquent d'éventuels recours, est sensiblement supérieur à celui des personnes placées en zone d'attente- il est d'environ 46 000 contre 8 000. Les cas d'appel d'une décision de fin de placement en zone d'attente sont donc plus exceptionnels que ce que l'on observe s'agissant des placements en centre de rétention administrative. Les conditions matérielles d'accueil et les droits des personnes maintenues en zone d'attente ou retenues en centre de rétention administrative diffèrent également. L'incidence d'un allongement de la durée de placement ne peut donc être considérée comme identique dans l'une et l'autre situation. situation. Les conditions de placement en zone d'attente sont d'ailleurs régulièrement critiquées, notamment pour manque de prise en compte du critère de vulnérabilité des personnes placées. Dans ces conditions, nous proposons la suppression de l'article 10 l'avis du rapporteur.

Le scrutin est ouvert.

Durain. Cet amendement vise à supprimer l'augmentation de six à dix heures de la durée pendant laquelle un étranger est maintenu à la disposition de la justice après notification mettant fin à son maintien en zone d'attente.

Le scrutin est ouvert.

Je considère néanmoins que, les conditions ne pouvant pas être réunies pour poursuivre ce

Monsieur le président Bas, avec tout le respect que je vous porte, je dois dire que, pour nous, les conditions de travail sont acceptables. Nous ne sommes pas responsables des manquements de certains groupes de la Haute Assemblée.

Le groupe que j'ai l'honneur de représenter, le groupe socialiste et républicain, est normalement présent dans cet hémicycle, après une mobilisation que nous avons souhaitée au regard de l'importance du texte qui nous est soumis.

mais qui, peut-être, seront majoritaires dans quelques instants, dans le cadre du rapport de force présent. Madame la présidente, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain souhaite continuer à travailler le temps qu'il faut pour que ce texte soit analysé dans les meilleures conditions parlementaires.

! Je pense que, pour les uns et pour les autres, il convient que nous ayons ce débat sur le fond. À l'heure qu'il est, nous connaissons une nouvelle crise en Méditerranée,

Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de maintenir des mineurs accompagnant leur famille en zone d'attente. L'enfermement des enfants en zone d'attente est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lequel « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération La privation de liberté pendant une durée pouvant atteindre vingt, voire vingt-six jours, avec le risque d'être réacheminé à tout moment, est par définition attentatoire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme relève que « la promiscuité, le stress, l'insécurité et l'environnement hostile que représentent [les centres de rétention] ont des conséquences néfastes sur les mineurs, contraires avec les principes internationaux de protection des enfants Cette décision est parfaitement transposable aux zones d'attente. Par ailleurs, la situation faite aux mineurs placés en zone d'attente est en contradiction flagrante avec le principe de protection des mineurs contre l'éloignement.

Unanimement, les salariés de la Croix-Rouge m'ont parlé des traumatismes que pouvait provoquer cette rétention des enfants, et de la frustration des familles qui ont des enfants en zone de rétention.

En juin 2015, le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, s'est saisi d'office de la situation de deux fillettes âgées de trois et six ans, retenues plusieurs jours dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy. À cette occasion, il a réaffirmé son opposition à l'enfermement des enfants en zone d'attente.

que le maintien en zone d'attente ne peut constituer qu'une mesure de dernier ressort et doit être d'une durée aussi brève que possible. Cela l'a conduit à formuler dix recommandations générales, afin de mieux garantir la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. cet amendement tend à l'interdiction générale et absolue de placer des mineurs en zone d'attente, dans la mesure où il s'agit d'une privation de liberté.

de ne pas être satisfaits de la manière dont ce débat se déroule. Les uns et les autres ! Pour autant, je crois que nous en avons suffisamment parlé et que la meilleure démonstration que de notre esprit de responsabilité, à nous tous qui sommes présents ce soir, est de continuer à travailler sur le fond, puisque la séance se poursuit, et de faire avancer le débat. La séance a

équivaudrait concrètement à devoir accepter l'entrée sur notre territoire de tout mineur isolé, de tout mineur, voire de toute personne accompagnée d'un mineur, du seul fait qu'ils se présentent à nos frontières.

des mineurs en zone d'attente est particulièrement encadré pour tenir compte de leur vulnérabilité. Outre les garanties reconnues à tout étranger, à savoir l'assistance d'un interprète et d'un médecin, la communication avec un conseil ou toute personne de son choix, le mineur bénéficie de protections spécifiques supplémentaires. En effet, doit être désigné pour le représenter dans le cadre de toutes les procédures administratives et juridictionnelles, s'il n'a pas de représentant légal. En outre, les conditions matérielles de maintien sont aménagées : il bénéficie ainsi, en pratique, à Orly ou à Roissy, d'un lieu d'hébergement adapté et séparé, que, comme beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, nous avons visité. Enfin, le réacheminement ne peut se faire qu'après s'être préalablement assuré de la prise en charge du mineur, soit par sa famille, soit par une institution chargée de le protéger.

je peux vous dire, en tant que ministre de l'intérieur, que nous connaissons un certain nombre de mineurs qui sont arrivés à Paris totalement asociaux.

Le problème des mineurs étrangers isolés présents sur notre territoire est une réalité, comme dans d'autres territoires en Europe. Il s'agit d'une réalité extrêmement forte. On a beaucoup parlé de Mayotte aujourd'hui. Et pourtant, des conventions internationales- parce que l'on croit à la protection de l'enfance -s'imposent à nous. J'espère que, au-delà des propos que vous avez tenus, votre idée n'est pas de renoncer à l'État de droit dans lequel nous sommes engagés, et qui fait l'honneur de la République, depuis 1789

! Ce qui nous sépare, monsieur le ministre, c'est que je ne fais pas de différence entre des mineurs asociaux français et étrangers : c'est ça l'humanité

dont on peut très bien deviner les origines, qui est issue de rapports que l'histoire ne cesse de dénoncer. Je ne comprends pas comment on peut traiter des enfants comme cela et les déshumaniser à ce point. Je ne comprends pas comment un peuple peut être traité de cette manière, surtout par le pays qui se dit le champion des droits de l'homme J'en suis très triste et, si je n'avais aucun motif de voter contre ce texte, ce moment précis m'en donne toutes les raisons ! Je suis très amer, monsieur le ministre.

nous faites faire un bond en arrière de trois siècles pour tenter de justifier les mesures complètement ahurissantes que vous souhaiteriez prendre en 2018

J'ai beau éplucher les dix-sept versets de cette religion laïque et obligatoire, je n'y ai pas trouvé l'obligation d'accueillir chez nous toute la misère du monde, même lorsqu'elle est mineure L'interprétation que vous en faites est purement idéologique et n'est absolument pas adaptée à la réalité de notre pays en 2018. Quelle bouillie ! Cela a été rappelé dans cet hémicycle, il y a quelques semaines, on estime que 70 % de ces mineurs, du moins déclarés comme tels,

une première mesure à prendre dans une démocratie responsable, surtout lorsqu'elle compte 9 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs : il faut obliger il faut obliger ces prétendus mineurs à accepter le test qui permet de déterminer si, oui ou non, ils sont mineurs et d'agir en conséquence. Mes chers collègues, il serait temps

L'honneur de la République, c'est d'aider ces enfants, qu'ils soient français ou étrangers. Le déshonneur, c'est d'ignorer leur souffrance et de les enfermer. Vous ne mesurez pas, monsieur le ministre d'État, les dégâts psychologiques produits sur un enfant, quel que soit le nombre d'heures pendant lesquelles il est privé de liberté. Le droit de l'enfant

la question des enfants, des mineurs, qu'ils soient isolés ou non, devrait faire consensus dans une enceinte républicaine ! Je dis bien une « enceinte républicaine ». Je

ailleurs, je m'étais fait une promesse en entrant dans cet hémicycle, voilà dix mois : ne jamais répondre à l'extrême droite. Sans cela, on lui donne

à une course à l'échalote. Vous courrez derrière l'extrême droite ! Vous légitimez les discours qui sont tenus, aujourd'hui, dans cet hémicycle ! C'est intolérable ! Pour la première fois, en France, un texte assimile asile et immigration. C'est un jeu très dangereux,

du dialogue, s'il s'agit d'un dialogue, on puisse s'emporter et franchir les limites, mais ce type d'accusations implicites est proprement intolérable. C'est Madame la présidente Assassi, je veux souligner à ce stade du débat, après tant de manifestations d'indignation, que la loi de la République n'a pas attendu le débat de ce soir pour se préoccuper de la situation des enfants étrangers qui arrivent dans nos aéroports. Je signale à nos collègues du groupe socialiste et républicain

ou des conditions supplémentaires au placement temporaire d'enfants étrangers dans les zones d'attente. Nous avons à trouver un bon équilibre entre plusieurs préoccupations. La préoccupation de la dignité de la prise en charge de ces enfants est évidemment un souci majeur, et croyez bien, mes chers collègues de la gauche, que ce souci est partagé sur toutes les travées. Les postures accusatoires sont tout à fait excessives et blessantes

? Les conditions d'accueil dans les zones d'attente obéissent à des prescriptions visant à assurer la qualité de l'environnement de l'enfant. On vous dit

qu'il peut être accueilli à son retour. Si bien que toute allusion à la barbarie nazie et aux camps de concentration est évidemment totalement déplacée, s'agissant de cette loi de la République que la gauche au pouvoir n'a pas cherché à modifier-

! Je crois qu'il est temps, ce soir, de revenir à une plus exacte appréciation de nos réalités et de notre droit. On peut fort bien refuser ces amendements, tout en ayant aussi

qui étaient tous, si j'ai bien compris, des tricheurs, des menteurs, des voyous, et des filles qui se préparaient à la prostitution. Cela

présentent constamment les immigrés- il faut écouter ce qui est dit, il faut penser à l'implicite -comme des tricheurs,

comment on considère l'ensemble des couches de la population, quelles sont mes relations- puisqu'on m'accuse de cela -avec

en Afrique pour porter une volonté de développement, lorsqu'il intervient auprès de l'Union européenne afin que des fonds pour le développement et pour la sécurité en Afrique soient octroyés, oui, nous menons une politique équilibrée

Le scrutin est ouvert.